complété par un nouvel alinéa, tendant à informer le consommateur en cas d'emploi de pesticides classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ces substances chimiques sont suspectées d'avoir un impact sur le dérèglement du système hormonal et de favoriser différentes maladies, comme l'obésité, le diabète de type 2, les troubles neurocomportementaux ou encore les cancers hormonodépendants. L'article 11 A, dans sa version initiale, a été supprimé en commission. Il est pourtant nécessaire d'informer le consommateur et de lui donner accès à l'ensemble des informations. savoir si, oui ou non, les denrées animales ou d'origine animale ont été nourries avec des organismes génétiquement modifiés et connaître le mode d'élevage, l'origine géographique, le nombre des traitements opérés sur les fruits et légumes ainsi que leur nature.

Si le bilan est positif, la mesure pourrait être étendue à l'ensemble des États membres. Poursuivons la même logique, et n'opposons pas nous-mêmes l'argument de la concurrence déloyale et des difficultés vis-à-vis du droit communautaire

aux États membres de l'Union européenne d'imposer des mentions complémentaires, si celles-ci se justifient notamment par des raisons de santé publique ou de répression des tromperies. N'attendons pas un prochain scandale sanitaire !

Une pétition, cosignée par plus de 30 000 de nos concitoyens, vient également soutenir cette disposition. Ainsi, l'étiquetage des denrées alimentaires est complété par un affichage environnemental comprenant d'une part, pour toutes les denrées animales ou d'origine animale, le mode d'élevage, l'origine géographique ainsi que, le cas échéant, pour les fruits et légumes frais, le nombre de traitements phytosanitaires. C'est une mesure de santé publique que nous devons à nos concitoyens. Par ailleurs, je rappelle que notre groupe, qui s'appelait anciennement « CRC », porte cette volonté d'étiquetage des denrées alimentaires depuis des années, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'OGM.

et pour les producteurs. Il est essentiel d'assurer l'information et la liberté de choix du consommateur, en garantissant un étiquetage clair. Les informations sur l'utilisation de produits phytosanitaires, sur le mode d'élevage et l'utilisation de produits OGM dans l'alimentation animale ou sur l'origine géographique ne sont que rarement disponibles. correspond pourtant à une demande croissante des consommateurs : toutes les études montrent que les Françaises et les Français se posent des questions sur leur alimentation. De même, de plus en plus d'agriculteurs adoptent des pratiques vertueuses, par exemple en ce qui concerne les bovins ou les vaches laitières élevées dans les systèmes herbagers : ils doivent pouvoir valoriser leur travail et la qualité de leurs produits par rapport à des systèmes fondés uniquement sur le maïs et le soja. Il faut valoriser, par un affichage clair, les pratiques vertueuses des producteurs. Cet amendement peut être compatible avec la réglementation européenne. Certes, le droit communautaire ne prévoit pas que les éléments cités à cet article fassent partie des informations communiquées aux consommateurs. En revanche, il prévoit qu'un État membre

supprimé en commission, qui prévoyait, à partir du 1 janvier 2023, certaines mentions obligatoires sur les denrées alimentaires mises sur le marché français. Toutefois, nous ne reprenons pas la mention relative au nombre de traitements par produits phytosanitaires sur les fruits et légumes, car, d'une part, nous nous interrogeons sur la faisabilité et la fiabilité d'un tel dispositif et, d'autre part, nous n'estimons pas souhaitable de cibler uniquement cette catégorie de produits. En outre, nous savons que la puissance des produits est au moins aussi importante aujourd'hui que le nombre de pulvérisations. Si étiquetage il devait y avoir sur les traitements phytosanitaires, il faudrait bien réfléchir aux modalités des mises en oeuvre, pour s'assurer que le consommateur dispose d'une information fiable et transparente. En tout état de cause, nous proposons la réintégration de l'affichage relatif aux OGM, au mode d'élevage ou encore à l'origine géographique des produits.

à avancer l'application à 2021 ou encore à ajouter la nature des traitements phytosanitaires sur les fruits et légumes. L'amendement n° 538 rectifié reprend la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exception du nombre de traitements rectifié ne vise que l'origine géographique pour les denrées d'origine animale. Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui a adopté six amendements identiques de suppression, satisfaisant par ailleurs trois amendements de suppression partielle. Je rappelle brièvement que les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées au niveau européen. Par conséquent, imposer des règles particulières en France soit pénaliserait nos agriculteurs, soit serait contraire à la libre circulation des biens si tous les produits commercialisés sur le territoire national étaient visés.

outre, certains signes d'identification de la qualité et de l'origine renseignent déjà sur le mode d'élevage. Enfin, le contrôle de cette obligation est impraticable, en particulier s'agissant du nombre de traitements phytosanitaires, qui, du reste, n'est pas un indicateur pertinent et desservirait notamment les produits bio. Pour toutes ces raisons, la commission émet

un an, nous avons obtenu de Bruxelles que la France puisse expérimenter l'étiquetage de la composition des aliments sous forme décroissante.

pour définir des règles très spécifiques de production ou de transformation qui apporteront encore plus de richesse et de valeur au produit.

portant sur la nature des traitements appliqués. Comme nous l'avons déjà souligné, il est temps de prendre en compte la forte demande sociétale exprimée lors des États généraux de l'alimentation et, plus largement, dans les différentes discussions que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, ce qui passe par une meilleure information des consommateurs quant à la qualité de leur alimentation. Enjeu public de premier ordre, la transparence sur la production des denrées alimentaires nous apparaît comme indispensable.

aux importations de soja génétiquement modifié dont la culture est interdite en France, mais dont l'importation est autorisée. En effet, bien qu'elle produise 55 % de ses protéines, la France est le plus gros importateur et consommateur européen de tourteaux de soja dont la majorité vient du Brésil- 22 % du soja exporté par le Brésil est destiné à la France. Cette mention permettra de créer une véritable dynamique en faveur d'une production d'alimentation animale 100 % française.

Une loi de la biologie a été violée, ce qui a entraîné l'apparition de maladies à prions. Le franchissement de la barrière des espèces, c'est un drame. Je veux bien que l'on défende tout et n'importe quoi avec n'importe quels arguments,

Monsieur Labbé,

Le scrutin est ouvert.

de mieux consommer, intégrant comme critère d'achat la notion de bien-être animal. Or les informations disponibles, relatives tant à l'élevage qu'au transport et qu'à l'abattage, ne leur permettent pas de mettre en pratique cette consommation responsable. Selon le dernier Eurobaromètre réalisé par la Commission européenne en 2016 sur l'attitude des Européens à l'égard du bien-être animal, 52 % des Français estiment estiment que l'offre des distributeurs en produits alimentaires respectueux du bien-être animal est insuffisante. Et comme en réponse, ils sont, selon la dernière étude ACCEPT réalisée par les instituts techniques des filières d'élevage, à 96 favorables à un étiquetage des produits selon le mode d'élevage- plein air ou non. D'où cet amendement dans lequel est proposée une expérimentation permettant de déterminer les conditions de mise en place de cet étiquetage.

l'information n'est pas toujours disponible et plusieurs études montrent que le consommateur est susceptible de mal interpréter les informations dont il dispose sur l'emballage.

valoriser ses produits et faire de la publicité d'une certaine manière mensongère. Il est donc nécessaire d'assurer un minimum de transparence. En outre, un tel étiquetage valoriserait les éleveurs, de plus en plus nombreux, qui, dès lors qu'ils pratiquent des modes d'élevage vertueux, méritent d'être encouragés. Ces modèles, s'ils sont valorisés auprès des consommateurs, sont plus rémunérateurs pour les éleveurs. Or tel est également l'objet de ce texte.

notion d'étiquetage obligatoire du mode d'élevage, mais l'étend au mode d'abattage et à tous les produits bruts ou transformés comportant des produits issus

: La parole est à Mme Angèle Préville. L'information environnementale obligatoire sur les produits alimentaires répond à une forte demande citoyenne, à un impératif de transparence des relations entre producteurs, distributeurs et consommateurs,

Pour répondre à la fois au besoin d'une information simple et courte et d'un affichage environnemental multicritères donnant une information juste et fiable, il est proposé d'articuler deux démarches : une information visible immédiatement en magasin et compréhensible par tous et une information plus exhaustive disponible en ligne. En ce qui concerne l'information relative à l'impact du dioxyde de carbone du produit, il est proposé de mettre la priorité sur la distance parcourue et le mode de transport. C'est la solution qui semble la plus pédagogique. À l'inverse, l'indication du nombre de grammes d'équivalent CO2 émis sur l'ensemble du cycle de vie du produit est est certes transparente, mais elle n'est pas pédagogique, puisqu'elle n'évoque rien pour la plupart des Français. Un format d'affichage très clair a été imaginé, qui pourra être transmis aux services de l'État en vue d'élaborer le futur modèle

Dans le cas de produits animaux, ces informations pourraient intégrer des éléments détaillés relatifs au mode d'élevage et d'abattage de l'animal. Les producteurs pourraient même être incités à fournir des photographies du lieu d'élevage des animaux, pour permettre au consommateur de constater par lui-même dans quel type de milieu les animaux sont élevés

excessivement contraignantes, par exemple l'indication de la distance parcourue du lieu de production jusqu'au lieu de distribution, qui serait du reste impossible à mettre en oeuvre puisqu'il faudrait autant d'étiquettes qu'il y a de lieux de distribution,

d'Amérique du Sud ou d'autres continents.

Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur et la transparence de la composition des plats préparés à base de minerai de viande. Le minerai de viande bovine est un produit intermédiaire constitué de muscles et de la graisse qui lui est attachée, issu de la découpe des carcasses et du désossage. Il est destiné à une transformation ultérieure, pour la fabrication de steaks hachés et de plats cuisinés. Le minerai étant un produit intermédiaire utilisé uniquement entre opérateurs de l'agroalimentaire, il n'est actuellement pas étiqueté sur le produit final remis au consommateur.

graisse. Rien ne justifie donc un étiquetage spécifique. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les steaks hachés ou les saucisses ne sont pas constitués d'autre chose que de minerai de viande. La commission est donc défavorable

Tissot. Cet amendement vise à encadrer certaines pratiques commerciales consistant à afficher des mentions valorisantes sur l'étiquette des produits, sans que le producteur en soit informé. Ce type de mentions crée une valeur, puisqu'elle donne le sentiment d'un produit de meilleure qualité, qu'il s'agisse d'un signe officiel de la qualité ou de l'origine ou d'une allégation portant sur le mode de production. Une note de 2017 du ministère de l'environnement fait ainsi apparaître que les consommateurs sont prêts à payer entre 5 % et 45 % plus cher pour un même produit ayant un moindre impact environnemental. Ainsi, 57 % des fruits et légumes produits en France pourraient porter la mention « zéro résidu de pesticides », puisqu'ils sont sous les seuils autorisés en cette matière. Dans le cas de produits résultant d'un tri des fruits et légumes, le recours à cette allégation environnementale peut aujourd'hui se faire sans que le producteur en soit informé. C'est également le cas pour l'utilisation des races bovines dans la valorisation des viandes et steaks hachés : un industriel peut trier parmi ses carcasses et utiliser la mention valorisante « viande charolaise », sans en informer le producteur. L'amendement vise donc à assurer un meilleur partage de la valeur : dès lors qu'une allégation valorise le produit, le producteur doit non seulement en être informé, mais aussi se voir restituer une partie de la valeur générée. L'encadrement de la valeur créée par ces allégations est un enjeu majeur de la transition agricole : tant que des allégations concernant le mode de production pourront porter sur des pratiques ne rémunérant pas les producteurs, la transition agricole vers des pratiques vertueuses restera bloquée.

pour y apposer une allégation, sans pour autant que le producteur soit rémunéré à hauteur de la valeur créée par ladite allégation.

du Gouvernement ? La répartition de la valeur au sein de la chaîne de production est un enjeu fort, de même que l'évolution des filières vers des modes de production responsables. Mais cela ne doit pas être encadré par des dispositions dont l'application serait excessivement coûteuse pour de nombreuses filières, ce qui pourrait freiner

sur l'opportunité de la mise en place d'un système de permettant de retracer la création de valeur d'un produit ou d'une denrée alimentaire sur l'ensemble de la chaîne de production, et de délivrer une information complète sur la composition des aliments transformés.

L'intérêt de la dans le domaine agroalimentaire, c'est de rendre complètement transparentes les données relatives aux produits commercialisés, de la ferme à la table du consommateur. Les données peuvent concerner la qualité nutritive des aliments et les modes de production. Elles peuvent aussi renseigner sur la répartition de la valeur économique tout au long de la chaîne, de la production à la commercialisation. À terme, les techniques de QR code sur smartphone permettront un accès généralisé à ce type d'information,

La création de valeur est déjà suivie et évaluée par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. C'est précisément l'objet des contrats et accords-cadres que de la retracer au travers des indicateurs qui sont prévus. Je suis par ailleurs assez sceptique quant à l'intérêt d'appliquer la théorie du à la création de valeur, qui ne renvoie ni à un problème de sécurisation des données ni à un enjeu de puissance de calcul disponible. Néanmoins, je vous propose de renvoyer ce sujet à l'OPECST,

Je ne voudrais pas que le monde agricole et agroalimentaire passe à côté de cette technologie. J'ai constaté sur le terrain que certaines entreprises en pointe mettaient en oeuvre ce type de technique, qu'il convient d'accompagner. Dans le cadre des plans de filière faisant suite aux États généraux de l'alimentation, le Gouvernement a prévu d'accompagner les filières dans leur modernisation.

Nos habitudes de consommation évoluent et internet devient un nouvel espace de consommation. Malgré ce changement d'usage, les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des mêmes exigences d'information et de transparence que dans le commerce traditionnel où le produit est palpable et l'étiquette, à portée des Les plateformes de vente en ligne de denrées alimentaires considèrent qu'elles remplissent leurs obligations d'étiquetage fixées par le code de la consommation et le règlement européen INCO en utilisant des photographies des produits. ce règlement prévoit que les informations obligatoires pour des denrées alimentaires doivent figurer sur le support de la vente à distance, ce qu'une simple photo peut satisfaire. En revanche, il n'impose aucune obligation quant à la transparence et au caractère explicite de ces informations : une photo de l'emballage n'est pas toujours directement apparente ni dans une police suffisamment lisible. lisible. L'article 11 , introduit avec le soutien du rapporteur à l'Assemblée nationale, prévoit une application fidèle du règlement INCO, dont les dispositions peuvent être aujourd'hui contournées par les plateformes. Une telle mesure vise à respecter le devoir d'information au consommateur.

visible de façon explicite. Une telle précision, ma chère collègue, est donc au mieux inutile, si elle ne fait qu'expliciter une règle déjà en vigueur. Elle pourrait même être non conforme au droit européen si elle

L'accessibilité en ligne de l'information sur les marchandises est, à terme, une des conditions de la transformation numérique de nos entreprises et de notre économie. Le secteur agroalimentaire est en première ligne de cette exigence d'accessibilité. En effet, la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande forte, constante et croissante des consommateurs, qui souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé et consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouvertes est la démonstration de l'intérêt des consommateurs. L'accès en masse à ces données est également indispensable à la recherche en matière de politique de santé publique et de nutrition. L'objectif de cet amendement est donc de poser le principe général de l'accessibilité en ligne des informations sur les marchandises et de définir par décret les conditions dans lesquelles le secteur agroalimentaire pourrait être le premier à à le mettre en application, dans des conditions relativement souples, et ce afin de soutenir notamment le développement d'applications mesurant la qualité nutritionnelle des aliments. Ainsi, le décret organisera la mise en des informations obligatoires d'étiquetage par les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires préemballées, à l'exception des TPE, en posant que ces informations devront être rendues accessibles sous format informatique ouvert et réutilisable dans des conditions non discriminatoires par tous. Le secteur agroalimentaire aura la charge d'organiser la mise à disposition de ces informations par les entreprises, dans des conditions harmonisées entre les filières. L'exclusion dans un premier temps des TPE du dispositif permettra d'en circonscrire l'obligation à des entreprises sachant déjà produire de la donnée structurée.

Tout ce qui est rendu obligatoire sur l'étiquetage, et uniquement cela, sera donc mis sur internet de manière claire et lisible. En revanche, la base ne serait pas ouverte, car il nous semble préférable de ne pas imposer de choix technologique par la loi. Notre amendement permet de poser le principe général de l'accessibilité en ligne des informations. Il reviendrait ensuite au secteur agroalimentaire de s'organiser pour la mise à disposition de ces informations par les entreprises, dans les conditions harmonisées par les filières. telle mesure répond au souhait des consommateurs de pouvoir effectuer un choix éclairé, afin de consommer mieux, plus durable et plus local. Elle favoriserait également l'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouvertes, de plus en plus utilisées par nos concitoyens.

ou PNNS, comme un axe d'articulation entre les deux. Là encore, il n'est pas nécessaire de passer par la loi. Mieux vaut encourager les professionnels dans les démarches qu'ils sont en train de mettre en place.

présenter l'amendement n° 147 rectifié. Cet amendement vise à encourager la mise en des informations d'étiquetage par le responsable des informations sur les denrées alimentaires, en permettant aux vendeurs de se référer à l'information que ce dernier aura partagée comme moyen de remplir les obligations de l'article 14 du règlement n° 1169/2011 sur la vente à distance. Il s'agit de permettre et de soutenir le développement d'applications autour de l'exploitation de ces données, mesurant la qualité nutritionnelle des aliments, mais aussi la mise en oeuvre de programmes de recherche- et intelligence artificielle -, autour de l'exploitation des informations sur les produits. Car la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs, qui souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé et consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données ouverts est la démonstration de l'intérêt des consommateurs.

ne souhaitent pas mettre en oeuvre le dispositif facultatif Nutri-score. L'exploitant aura le choix et l'occasion de mettre en ses informations produit pour que des tiers structurent et présentent ces données à leur place. Il s'agit de renforcer la transparence et d'utiliser les possibilités offertes par le numérique à notre avantage.

prévoient l'obligation, pour les « exploitants du secteur alimentaire », dont on imagine qu'il s'agit des producteurs, de mettre l'ensemble des informations sur les « denrées alimentaires », là encore sans plus de précision, en.

C'est exactement la question qui s'est posée pour les fromages fermiers. Un fromage est-il fermier parce qu'il est fabriqué et affiné en totalité à la ferme ? Les cas sont tout de même très limités. Ou bien peut-il être affiné ailleurs et bénéficier néanmoins de ce label de qualité ? Il faut répondre à cette question juridique. Le texte, me semble-t-il, y répond. Oui, un fromage peut être fermier avec un affinage en dehors de la ferme, sous réserve du respect de méthodes d'affinage traditionnelles, d'une part, et d'en informer le consommateur sur l'étiquetage du fromage, d'autre part ! Cet article permet de sécuriser les producteurs qui affinent leurs fromages en dehors de la ferme et qui pratiquent déjà l'étiquetage avec la mention explicite

instiller des peurs sur de tels sujets. Nous ne remettons pas en cause ce qu'est un fromage fermier. Nous encadrons les usages, en conformité avec des cahiers des charges qui sont compliqués à tenir et rigoureux, mais qui permettent de bien valoriser les productions issues des productions fermières.

Cet amendement tend à supprimer l'article 11 , relatif à l'ouverture de la dénomination « fromage fermier ». Cet article introduit une nouvelle définition du fromage fermier en admettant la possibilité d'un affinage en dehors de l'exploitation agricole. Or la mention valorisante « fermier » est définie par le décret n° 2007-628 et se limite aux fromages « fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci Dans la nouvelle disposition, l'association des notions « fromages fermiers » et « affinage hors de l'exploitation » pose problème aux producteurs laitiers fermiers à plusieurs titres. Tout d'abord, lorsque le processus qui va du lait au produit fini affiné est réalisé entièrement sur une même ferme, l'identité du producteur et la provenance du produit sont clairement connus du consommateur l'étiquette. C'est évident. Toutefois, lorsque l'étape finale d'affinage a lieu hors de la ferme, c'est souvent la marque, donc l'identité du seul affineur qui est mise en avant. Là, c'est très fréquent ; affineur, c'est un vrai métier. Cela induit, d'une part, une perte de traçabilité pour le consommateur, qui aura du mal à savoir où et comment le produit concerné a été fabriqué, et, d'autre part, une perte de valeur ajoutée pour le producteur fermier, alors même que c'est son travail qui rend possible l'utilisation de la mention valorisante « fermier » sur le produit. Enfin, il faut le noter, l'introduction d'une telle disposition va à l'encontre d'une décision du Conseil d'État, qui a fait supprimer la possibilité d'affinage des fromages fermiers à l'extérieur de la ferme, en se fondant sur les arguments selon lesquels l'affinage est partie intégrante de la fabrication d'un fromage affiné. Le producteur agricole doit être directement responsable et les pratiques d'affinage doivent être traditionnelles.

Il considère que nous risquons d'envoyer un message brouillé au consommateur et une dilution de la traçabilité, l'identité de l'affineur occultant celle du producteur.

tout en assurant une bonne information des consommateurs, dès lors qu'il sera indiqué de manière claire et précise que l'affinage a eu lieu en dehors de la ferme. Le consommateur pourra donc choisir en toute connaissance entre un fromage fermier affiné à la ferme et un fromage fermier affiné en

pour explication de vote. Notre amendement est soutenu par l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers, qui représente 16 organisations et regroupe 914 producteurs adhérents.

La suppression de l'article va donc, me semble-t-il, dans l'intérêt des 6 000 producteurs laitiers fermiers, qui, pour la grande majorité, affinent eux-mêmes leurs fromages et dont l'efficacité économique dépend essentiellement de la plus-value jusqu'à présent attachée à la mention

au droit actuel, qui n'offre pas du tout de cadre juridique sécurisé pour les producteurs, pas même pour ceux qui sont en zone AOP. D'ailleurs, monsieur le ministre, en écho à votre invitation, je pense qu'il serait

Et il est très important de le dire : combien de producteurs fermiers disparaîtraient si on ne leur permettait plus d'affiner collectivement les fromages fermiers qu'ils produisent en plus de ceux qu'ils vendent directement ? Car c'est ça la réalité !

est affiné ailleurs, on précise où et par qui. Au moins, il y a une très grande transparence. Merci de cet amendement, qui vraiment sécurise le système fermier de notre pays

égard aux arguments de Mme le rapporteur et de M. le ministre, nous retirons notre amendement.

très peu de saint-nectaire peuvent être affinés à la ferme. Il s'agit pourtant bien d'un fromage fermier qui respecte les traditions, et la position de l'Assemblée nationale a été très claire : on marque bien qui affine et on précise « dans les conditions traditionnelles

de l'article pénalise fortement les producteurs fermiers, qui ne pourront plus faire valoir leur travail. Elle pénalise aussi les consommateurs, qui ne pourront plus identifier clairement les produits. L'amendement vise à prévoir que le

Il est la transposition d'une pétition signée par plus de 35 000 personnes, dont les grands chefs Antonin Bonnet, Michel Bras et William Frachot, qui vous a été remise mardi, monsieur le ministre. L'article 11, dans sa rédaction actuelle, ouvre la voie à une confusion. Sa simple suppression, cela a été dit, ne suffit pas ; nous ne la souhaitions d'ailleurs pas. Aujourd'hui, l'appellation « fromage fermier » est strictement encadrée. Pour obtenir cette appellation, un fromage doit être produit et affiné dans la ferme du producteur. Si l'article est voté tel quel, demain, un fromage affiné en dehors de la ferme pourra être appelé « fermier » sans autres contraintes. Nous risquons donc d'entraîner une confusion dans les produits et en conséquence de léser des producteurs. Cela pourrait s'accompagner d'une perte de qualité pour des raisons lucratives, peu respectueuses de nos savoir-faire et du travail paysan.

C'est nos savoir-faire et nos artisans qui sont en danger. Aussi, contrairement à l'essentiel des amendements en discussion commune sur cet article, nous demandons que l'étiquetage précise le nom du producteur. Sinon, c'est l'authenticité d'un travail qui risque de se perdre. Nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement plein de bon sens et pragmatique pour préserver la richesse et la diversité de nos produits.

Le scrutin est ouvert.

: La parole est à M. François Bonhomme. La valorisation des produits de qualité et de tradition constitue un élément d'identification et de commercialisation important pour nos territoires ; cela se traduit souvent par une dénomination courante qui peut contribuer fortement à sa notoriété. Le présent amendement vise compléter l'article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime qui vise à définir les objectifs de la « politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer en précisant que la valorisation du nom d'usage et de notoriété d'un produit répond à un de ces objectifs importants. La valorisation d'un produit implique une origine, une fabrication locale, une qualité contrôlée, un savoir-faire préservé et une notoriété dûment établie. Cet amendement permettra ainsi de reconnaître cette singularité. Une telle évolution sera de nature à redonner leurs lettres de noblesse à de nombreux produits locaux. Ce sera, par exemple, le cas d'une viennoiserie dont historiquement le nom a puisé son origine dans la région Gasconne et qui fait la fierté de tout le sud de la France, je veux bien évidemment parler de la chocolatine, et non du pain au chocolat.

comme une valorisation d'appellation d'usage courant parmi les objectifs de la politique promouvant la qualité et l'origine des produits alimentaires. Nous sommes bien évidemment tous, mes chers collègues, attachés à nos multiples appellations régionales, mais est-il vraiment nécessaire d'ajouter de telles précisions

s'appelle chocolatine dans le sud ou pain au chocolat comme c'est le cas chez moi, dans le Cotentin, peu importe

de plus en plus nombreux, qui transforment en farine les céréales de leur exploitation sont actuellement soumis à la même réglementation que les meuniers, ce qui entraîne des obligations spécifiques, notamment des règles sanitaires lourdes davantage adaptées aux productions industrielles. Ces agriculteurs ne sont pas meuniers, mais bien agriculteurs : ils font oeuvre de diversification. Leur activité de mouture est une activité agricole à part entière puisqu'il s'agit d'une transformation de leur propre production. Il est donc absurde et anormal qu'ils soient soumis aux normes et contrôles de la filière meunière. Ces normes sont en décalage complet avec la réalité de leur activité. Elles ont été élaborées pour des volumes considérables, avec une multiplicité d'opérateurs et une diversité d'origine des matières premières des filières industrielles. Cet amendement vise donc à clarifier le statut de ces agriculteurs et à alléger les normes auxquelles ils sont soumis, en marquant une distinction claire avec le statut de meunier.

l'amendement vise à fonder la distinction entre activité agricole et activité de meunerie sur le seuil défini par le décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, soit 350 quintaux de blé tendre par an.

Mes chers collègues, dès lors qu'un agriculteur possède et utilise un moulin, il n'y a pas lieu de l'exonérer des règles applicables en la matière, sachant toutefois que l'article L. 666-6 du code rural exonère déjà

clairement préciser dans la législation que la mention du pays d'origine doit figurer de manière évidente sur les étiquettes des bouteilles de vin. Il s'agit d'éviter les tromperies, d'éviter que ne soient induits en erreur les consommateurs. Quelle est la situation actuelle ? Les vins espagnols par exemple, pour ne citer qu'eux, sont présentés dans les rayons de manière dissimulée, déguisée ou maquillée, avec pour objectif de rendre méconnaissable ou inapparente leur origine.

Or tel n'est pas très souvent le cas. En commission, j'ai cité le cas de ces bouteilles de vin espagnol qui affichaient ostensiblement sur leurs étiquettes la cité de Carcassonne. N'y a-t-il pas là tromperie ? Très souvent aussi, l'origine de ces vins est rendue volontairement inapparente. N'y a-t-il pas là duperie ? La profession qualifie, à juste raison, ces pratiques de concurrence parasitaire, car elles n'ont d'autre but que de détourner au profit des vins étrangers l'image et la renommée des vins français pour mieux en récupérer la valeur économique. Faut-il laisser les choses perdurer ? On me dit que le droit européen répond au problème que j'expose et que les mesures à prendre relèvent, par ailleurs, du domaine réglementaire. Or, mes chers collègues, si l'une ou l'autre de ces réponses avait une quelconque efficacité

Or ces duperies et pratiques déloyales perdurent dans l'indifférence de tous, au détriment de nos filières viticoles. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter le présent amendement.

sont préjudiciables à toute une filière, laquelle est importante puisqu'elle représente 15 % de la production agricole française. La clarification des règles d'étiquetage par l'indication visible de la provenance de ces vins est donc primordiale pour assurer l'information claire et loyale du consommateur sur la provenance des produits et pour soutenir cette filière en mettant fin à cette concurrence déloyale. Pour ces raisons, nous vous demandons de réintroduire cet article, qui renforce notre législation en prévoyant que

On nous dit que le droit européen est censé régler ce problème. Or, sur le terrain, il ne règle rien du tout.

et donc efficaces, décident de s'emparer du problème et de proposer d'inscrire dans la loi les dispositions qui font défaut aujourd'hui.

Je voudrais mettre le doigt sur deux points. Tout d'abord, les moyens que l'État français consacre, ou entend consacrer, aux contrôles

et d'extension de l'étiquetage, notamment pour les produits viticoles.

Le scrutin est ouvert.

les raisins peuvent être importés dans un pays, vinifiés dans un autre et prendre l'appellation du pays où ils ont été vinifiés. Afin que ce soit plus clair pour les consommateurs, nous demandons que soit bien mentionnée l'origine

Si cette formulation était adaptée au contexte de l'époque, elle était depuis devenue source de contraintes et une entrave au développement de nouvelles productions. C'est pourquoi

de décembre 1957, qui va permettre une évolution de la production de la Clairette de Die et du Crémant de Die. Les producteurs pourront ainsi déposer de nouveau un cahier des charges pour l'AOC Clairette de Die

importés étant bien inférieurs, cet amendement prévoit que l'origine géographique des spiritueux vendus par les professionnels de la restauration soit mentionnée de façon lisible sur les cartes présentées aux consommateurs, comme cet article le prévoit pour l'origine des vins. Le

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux vous parler du miel. L'image de cet aliment est particulièrement positive dans l'opinion puisqu'on prête au produit du patient travail des abeilles ouvrières de nombreuses vertus, du point de vue tant gustatif que sanitaire. Nous sommes l'un des pays les plus réputés pour la qualité et la variété de ses miels, qu'ils soient produits dans les plaines du Gâtinais, dans les collines de la Drôme, dans les hauteurs du Trièves ou dans les forêts profondes de Bigorre. Le problème, c'est que la grande distribution faisant de tout produit une simple course à la rentabilité a tenté d'imposer une sorte de « miel standard produit de mélange de miels de provenances diverses. Or le miel a une signature, comme ce peut être le cas pour un bon vin ou un fromage- nous venons d'en parler miel de sapin, ce n'est pas pareil que le miel de chêne ou le miel de framboisier ou d'arbousier. Le miel, c'est un peu la nature qui vient en témoignage. C'est la signature de la biodiversité, comme le montrent désormais les « miels urbains » récoltés dans nos villes de banlieue ou dans la capitale, qui tirent parti de la grande variété des plantations effectuées en ville. Apiculteur est un vrai métier, à l'égal de vigneron ou d'éleveur laitier fabricant de fromages. Cela doit se respecter. Il est donc logique que l'étiquetage du miel soit précis et ne permette pas de leurrer le consommateur quant à la qualité du produit proposé. Je suis saisi

s'agit de rendre obligatoire un ordre d'étiquetage selon l'importance de la part prise dans la composition des mélanges de miels. C'est exactement le même

L'indication des pays d'origine dans l'ordre d'importance tient compte à la fois de la variabilité des approvisionnements et de la nécessité d'informer correctement le consommateur sur l'origine des miels en cas de mélange. À défaut de cette précision, et donc avec uniquement l'affichage de la liste des pays d'origine, des conditionneurs pourraient tout à fait induire le consommateur en erreur en mettant par exemple la France en premier, alors que les produits d'origine française ne contribueraient que pour une part très faible au mélange. Cette obligation nouvelle s'accompagne par ailleurs d'un report au 1 septembre 2020 de la date d'entrée en vigueur, de manière à laisser davantage de temps aux conditionneurs pour s'adapter à ces nouvelles exigences d'affichage. L'avis est donc défavorable.

Il est contradictoire d'être, à la fois, pour la rédaction adoptée par les députés et contre la rédaction adoptée en commission par le Sénat sur le même fondement.

Je vous rappelle que la France a obtenu que l'on expérimente l'étiquetage avec l'ordre décroissant. Si on peut le faire pour le reste, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour le miel ?

Mme la rapporteur. J'apporterai juste une précision. Objectivement, à partir du moment où il y a mention de tous les pays d'origine, il y a surtransposition. Ce que propose la commission, c'est d'aller au bout de la démarche et d'identifier d'où viennent ces miels.

Le code de la consommation définit déjà comme pratique commerciale trompeuse toute pratique reposant sur les « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur [ ...] les caractéristiques essentielles du bien ou du service [dont] son origine ». Mon cher collègue, l'usage du drapeau tricolore ou de la carte de France entre très clairement

tirer les enseignements de l'expérimentation qui est en cours. L'expérimentation que nous avions obtenue de l'Union européenne se fera d'ici à la fin de l'année. Cette évaluation nous servira bien évidemment à progresser

par des affichages ou par défaut d'information précise. Chaque fois que l'on peut aller dans le sens d'une meilleure information du consommateur, on va dans le bon sens ! Cet amendement, cosigné par de nombreux sénateurs de tous bords, vise à indiquer le lieu de production des matières premières utilisées sur l'étiquette des produits alimentaires transformés. Pour les produits bruts, cette disposition existe déjà. Par exemple, le consommateur est libre de choisir des fraises espagnoles ou des fraises françaises. Pour les produits transformés, il s'agirait d'inscrire le lieu de production des principaux ingrédients. Le consommateur doit pouvoir être en mesure de connaître dans quelle partie du monde est produite son alimentation. Cela éviterait des scandales, comme celui des sauces italiennes produites avec des tomates chinoises, certaines sauces étant même étiquetées en bio ! Cette disposition permettrait aussi d'être beaucoup plus transparent sur la traçabilité et l'aspect sanitaire des aliments.

qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. Ainsi, cet amendement semble répondre parfaitement à cet objectif européen et permettrait d'apporter aux consommateurs une information qu'ils sont en droit d'avoir.

va bien au-delà de ce qu'exige effectivement- cela a été évoqué -le droit européen. Il nous semble essentiel que ce type de démarche soit négocié, monsieur le ministre, et harmonisé au niveau européen.

amendement. On nous dit à chaque fois « l'Europe » et « il faut attendre ». Là, il y a urgence à ne plus attendre ! On l'a évoqué dans le cadre de la restauration collective : les 80 % de viande bovine

de très bons sens, qui sera très bien perçu. Alors si ça dérange un peu les opérateurs, eh bien ils iront s'approvisionner en viande française, tout simplement ! On cessera d'aller dans le plus bas de gamme, en dessous de tout ... Je mets aux voix